Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, c’est avec tristesse que nous avons appris, le 25 novembre dernier, la disparition de Gérard Collomb. Gérard Collomb nous a quittés au terme d’un combat contre la maladie, qu’il menait avec un grand courage. Ce matin même, ses obsèques se sont déroulées en la cathédrale Saint Jean de Lyon, en présence du Président de la République et de Mme la Première ministre, qui va nous rejoindre. Lors de cette cérémonie d’adieux, à laquelle assistaient de nombreux habitants de sa ville et de son département, ainsi que de nombreuses personnalités politiques, l’émotion était, je le sais, présente. Mathieu Darnaud, notre premier vice président, y représentait le Sénat. Figure emblématique de la capitale des Gaules, Gérard Collomb voua sa vie entière à un engagement inlassable au service de ses compatriotes et de l’intérêt général. Ses facultés d’écoute, son esprit de solidarité étaient unanimement salués et suscitaient le respect. Son élection, en 2001, à la mairie de Lyon restera le moment privilégié de sa vie publique. Il se consacrera à sa ville durant plus de dix sept ans. Grâce à lui, Lyon fut capable de rivaliser avec les autres métropoles françaises et européennes, sans pour autant perdre son âme. Il transformera sa ville et mettra toute son énergie au service de ses habitants ; énergie qu’il mettra aussi au service de la communauté urbaine de Lyon, dont il fut le président. fut aussi parlementaire, élu député dans la deuxième circonscription du Rhône, en juin 1981 ; il avait 34 ans. Son arrivée au Sénat, en novembre 1999, marquera sa vie politique. Il sera réélu en 2004 et en 2014. Il siégea au sein du groupe socialiste, alors présidé par Claude Estier. Il devint membre de la commission des affaires culturelles. Toujours tourné vers la modernité, il est, en 2007, l’auteur d’une proposition de loi relative à la coopération internationale des collectivités territoriales dans le domaine des technologies de l’information et des communications. En 2009, il intégra la commission des lois, où ses collègues d’alors peuvent témoigner de sa connaissance des dossiers touchant aux collectivités territoriales et à la décentralisation. le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, en juin 2013, à propos des compétences de la métropole de Lyon ; ce fut, je le sais, un temps majeur de sa vie de sénateur. Après avoir été l’un des principaux soutiens d’Emmanuel Macron, il est nommé ministre d’État, ministre de l’intérieur, dans le gouvernement d’Édouard Philippe. Il porte alors devant le Sénat le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, visant à transposer dans le droit commun certaines mesures de l’état d’urgence, et défend, en 2018, le projet de loi sur l’asile et l’immigration. Il doit affronter l’attentat islamiste de Trèbes et mesure le danger du communautarisme qui ronge notre pays. Lors de son départ du ministère de l’intérieur, il laisse ce message : « Aujourd’hui, on vit côte à côte ; je crains que, demain, on ne vive face à face. » C’est à méditer. L’hommage que nous lui rendons aujourd’hui n’est pas uniquement solennel. C’est un hommage à un humaniste, un hommage à un défenseur inlassable de sa ville de Lyon et de la métropole. À ses anciens collègues, j’exprime notre sympathie. À son épouse, à qui j’ai écrit, à ses enfants, à toute sa famille et à tous ceux qui ont partagé ses engagements, je souhaite redire la part que le Sénat prend à leur chagrin. Je vous propose d’observer un instant de recueillement.

Je veux remercier

ce matin, autour de sa famille et de ses proches, autour du Président de la République, autour des habitants de sa ville, nous avons dit adieu à un grand républicain, à un Lyonnais passionné et à un homme d’État. Gérard Collomb était un modèle de réussite républicaine. Rien ne le prédestinait ni à diriger sa ville ni à occuper d’éminentes fonctions ministérielles. Pourtant, sa passion pour les lettres, sa force de travail et la puissance de ses convictions lui ont permis de devenir enseignant, député, sénateur, ministre d’État, ministre de l’intérieur et, bien sûr, maire. Gérard Collomb a été l’homme d’une ville. Pour Lyon, il avait un amour réel, sincère, inébranlable. Arpenter sa ville, c’est croiser à chaque coin de rue ses projets, ses idées, ses intuitions. Il s’est donné corps et âme à sa ville et l’a transformée. Les Lyonnais ne l’oublieront jamais. Gérard Collomb, c’était encore un homme de conviction, porté par la volonté de servir au delà des clivages, porté par l’attention aux problèmes des Français plutôt qu’aux étiquettes politiques. Le Sénat, chambre des territoires et de l’apaisement, lui correspondait bien, et chacun dans la majorité présidentielle sait ce qu’il lui doit. doit. « » – vers les voies célestes par des chemins étroits – était une de ses devises. Aujourd’hui, Gérard Collomb a rejoint ces voies célestes, mais son empreinte restera. Il a changé la vie des Lyonnais. Il a changé la vie des Français. L’ordre

Leur libération est un premier pas, qui suscite un immense soulagement. En premier lieu, madame la ministre, pouvez vous nous informer sur l’état de santé de ces enfants, âgés de 12 à 16 ans, après des semaines de captivité ? je voudrais rappeler que, parmi les 1 200 civils tués lors des attaques du 7 octobre, 40 d’entre eux possédaient la nationalité française. Nous ne devons pas oublier nos compatriotes assassinés.

À ce sujet, je tiens à rendre hommage aux agents de notre corps diplomatique, qui travaillent d’arrache pied avec leurs collègues d’autres pays pour obtenir la libération des otages encore captifs. Madame la ministre, disposez vous de renseignements à leur sujet, pouvez vous nous donner de leurs nouvelles ? Enfin, la trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée jusqu’au 30 novembre. Il est permis d’espérer que ce soit un signe favorable à une désescalade, que vous avez publiquement appelée de vos vœux, même si nous n’ignorons pas que les négociations sont très difficiles. Madame la ministre, que pouvez vous nous dire de ces discussions et des perspectives qu’elles ouvrent ? La parole

de nos compatriotes retenus en otage est la priorité numéro un du Président de la République et de notre diplomatie. Je veux remercier de nouveau, comme le Président de la République et la Première ministre l’ont fait, tous ceux qui ont œuvré pour cette libération. Je pense en particulier au Qatar, à Israël, bien sûr, et à l’Égypte. Jour après jour, croyez le, nous avons été actifs et mobilisés, comme eux, pour obtenir ce résultat. Je vous remercie d’ailleurs de ce que vous avez dit à propos de nos agents diplomatiques et consulaires. Nous avons partagé parfois, souvent, l’inquiétude des familles. Aujourd’hui, nous partageons leur joie. Mais c’est aussi une joie mêlée de douleur, en pensant à ce que ces enfants ont vécu, en sachant que, s’ils sont désormais en sécurité et avec leurs familles, ce qui leur est arrivé est proprement inhumain. Cela doit nous rappeler quelle est la vraie nature du Hamas : une organisation terroriste et dénuée de tout scrupule. scrupule. Nous poursuivons nos efforts, tous nos efforts, sous la conduite du Président de la République, et nous restons pleinement mobilisés pour obtenir la libération de tous nos compatriotes retenus en otage. Nous ne relâcherons pas nos efforts, vous le savez, car la France n’abandonne jamais les siens.

À sa famille, à ses amis, à tous ceux qui l’ont connu et aimé, les sénateurs de mon groupe adressent leurs plus sincères condoléances. Sa disparition est une tragédie. Il est tentant, dans ces moments là, de céder à la colère, à la peur et à la division. Il est tentant de chercher des boucs émissaires, de stigmatiser, mais c’est précisément ce que veulent ceux qui cherchent à nous opposer les uns aux autres : tous ceux qui ont pour seul horizon la division. Rapidement, l’extrême droite a instrumentalisé l’affaire de Crépol. Et une ultradroite décomplexée a pris le relais dans les rues de plusieurs villes de France. Madame la secrétaire d’État, avec 1 300 fichés S, ces groupuscules représentent la deuxième menace terroriste en France. Il faut que tous nos concitoyens mesurent ce danger. ce danger. Les dissolutions de milices ne suffiront pas au combat contre la haine. Ces milices renaissent de leurs cendres, car les idées restent. C’est donc aussi la bataille des idées qui éloignera notre pays du risque de batailles rangées. Restons vigilants et déterminés. Aidons les jeunes de tous les territoires à se réapproprier les principes républicains, un axe qu’a porté ici le RDSE la semaine dernière lors de l’examen de son texte sur la citoyenneté. Nous devons aussi avoir confiance en la justice, en ses représentants et en sa capacité à maintenir la paix sociale. Dans un État de droit, c’est la justice qui doit rendre la justice. Madame la secrétaire d’État, une certaine catégorie de la classe politique a soufflé sur les braises de la violence. Il y a urgence à agir. Nous vous demandons de condamner, sans équivoque, les discours de haine et de division. Nous avons un devoir d’unité face à une société fragmentée, où le lien social est rompu, où le vivre ensemble est sérieusement menacé par toutes les minorités violentes. Madame la secrétaire d’État, comment comptez vous empêcher les prochaines expéditions envisagées par l’ultradroite ? La

Monsieur le sénateur Ahmed Laouedj, je vous remercie infiniment de votre question et d’avoir eu un mot pour le jeune Thomas. Tous les mots que nous pourrons prononcer les uns et les autres ne seront jamais à la hauteur d’une telle perte, pour ses parents et pour le pays.

profondément. Nous ne cesserons de le répéter, nous condamnons avec la plus grande fermeté les groupuscules d’extrême droite, qui prétendent se substituer aux policiers ou aux gendarmes pour se faire justice eux mêmes. Je vous l’assure, la réponse de l’État sera implacable face à ces porteurs de haine, qui ne cherchent qu’à nous diviser. Nous n’hésiterons pas à dissoudre des associations et groupuscules d’extrême droite, s’il le faut, comme nous l’avons toujours fait, avec Génération identitaire, par exemple. Le ministre de l’intérieur et des outre mer proposera notamment, lors du prochain conseil des ministres, la dissolution de la Division Martel, ce groupuscule infâme. Les forces de l’ordre sont également pleinement mobilisées pour interpeller les auteurs de ces troubles à l’ordre public, les traduire devant la justice et prévenir de nouvelles actions violentes. À Romans sur Isère comme à Lyon, de nombreuses interpellations ont eu lieu pour mettre fin à ces manifestations sauvages qui ne véhiculent que la haine de l’autre. Je rappelle également que treize attentats d’ultradroite ont été déjoués depuis 2017 par nos services de renseignement. Vous le voyez, monsieur le sénateur, l’État ne transige pas avec ce sujet gravissime pour la désunion de notre nation.

Mort aux bougnoules » : c’est avec ces trois mots peints sur le portail de la mosquée que les habitants de Cherbourg en Cotentin se sont réveillés samedi dernier. Ces menaces de mort sont intolérables. Ces mots sont abjects et d’une grande violence. Ils ont suscité un émoi légitime dans notre ville, peu habituée aux expressions de haine. Je reprendrai les mots de l’un des fidèles de la mosquée : « En écrivant cela, ils nous menacent physiquement, mais ils cherchent aussi à nous exclure de la communauté nationale. En effet, au travers de ces menaces, c’est bien notre communauté nationale, dans son entièreté, qui est touchée et meurtrie. Hélas ! les actes vécus samedi dans la Manche ne sont pas isolés. Dès le printemps dernier, notre collègue Jérôme Durain alertait et proposait une résolution dénonçant les violences commises par l’ultradroite. Depuis des mois, ces violences se multiplient partout dans notre pays : à Saint Brieuc, à Saint Brevin les Pins et dans bien d’autres lieux encore. Pas plus tard qu’hier, ce sont des croix gammées qui ont été découvertes sur la façade de la mairie de Lunas, dans l’Hérault. Depuis la mort tragique du jeune Thomas, à Crépol, nous constatons une recrudescence de ces actes. Des individus peu scrupuleux utilisent un drame qui nous atteint toutes et tous pour mettre à exécution leur obsession d’une guerre civile et ethnique. Dans ce climat de grande tension, nous déplorons sincèrement que le chef d’un grand parti républicain se refuse à condamner l’expédition punitive menée à Romans sur Isère par des militants d’ultradroite. Nous devons prendre la pleine mesure de notre responsabilité historique. Quand la cohésion nationale se fissure sous les saillies d’une violence débridée, quand la concorde républicaine est menacée par les défilés de groupuscules fascisants, aucun républicain sincère ne doit manquer à l’appel. Nous devons plus que jamais veiller à préserver la fraternité républicaine devant la recrudescence des actes racistes, antisémites et antimusulmans, qui menacent notre unité. Madame la secrétaire d’État, comment comptez vous faire front contre la haine et restaurer l’ordre républicain face aux menaces et aux violences de l’ultradroite ?

Je veux affirmer mon plein soutien et celui de l’État à nos compatriotes de confession musulmane de ce département, touchés par ces actes odieux. Ces croix celtiques qui ont notamment été taguées sont le symbole emblématique, comme vous le savez, de l’ultradroite. En ce sens, j’entends votre inquiétude légitime, inquiétude légitime, mais soyez rassuré : la République est et sera toujours intransigeante avec ces milices. Comme l’a précisé le ministre de l’intérieur et des outre mer, une enquête est en cours et les forces de l’ordre sont d’ores et déjà à pied d’œuvre depuis ce week end pour retrouver les auteurs de ces dégradations racistes, parce qu’il faut dire les mots, afin qu’ils puissent être présentés devant la justice. Monsieur le sénateur, vous le savez, le respect de toutes les croyances est inscrit à l’article premier de notre Constitution et s’impose à tous. Jamais nous ne laisserons ces mouvances d’ultradroite piétiner notre cohésion nationale. Nous n’abandonnerons pas nos compatriotes de confession musulmane qui vivent sereinement leur foi dans le respect des valeurs de la République. Je ne me résignerai jamais, nous ne céderons jamais

La République leur fera face partout où ces derniers sèmeront leur idéologie mortifère, infâme et, encore une fois, d’un autre âge. La parole

créé chez les Français une profonde émotion, une émotion sincère, une émotion légitime. Nous avons aussi vu, dans les minutes qui ont suivi, alors que le sang de Thomas était encore chaud,… Ça va bien ! … une ignoble tentative d’instrumentalisation organisée par l’extrême droite, qui s’est livrée à un racolage électoral répugnant. Nous avons entendu Mme Maréchal Le Pen parler d’une « guerre ethnique ». Nous avons entendu M. Zemmour parler d’une « guerre de civilisation Nous avons entendu Marine Le Pen parler des « petits blancs contre les personnes de couleur ». Ce sont les mots employés. Ensuite, il y a eu les actes, ces événements dans le quartier populaire de Romans sur Isère, avec des individus cagoulés, armés de barres de fer, qui étaient là pour casser du noir et de l’arabe. Ceux qui appartiennent à ces

Vous nous avez annoncé, et c’est tant mieux, la dissolution d’un certain nombre de groupes d’extrême droite. Nous nous en félicitons. Il reste que, derrière, il y a des donneurs d’ordre qui ont micro ouvert sur un certain nombre de chaînes de télévision pour répandre leur bile raciste. C’est la raison pour laquelle je vous demande, madame la secrétaire d’État, quand le Gouvernement va se saisir de la proposition de résolution des parlementaires communistes qui vise à rendre inéligibles les auteurs de propos racistes et antisémites ? Il est grand temps

Vous avez raison, l’ultradroite est un danger, un danger permanent contre la République et les valeurs universelles qu’elle porte en elle. Nous devons tous, unanimement, condamner avec la plus grande fermeté ces groupuscules identitaires, qui ne cherchent qu’une chose : l’affrontement. Les Irlandais ont pu notamment en constater les dégâts et la dangerosité ces derniers jours. En ce sens, monsieur le sénateur, nous n’avons pas attendu les récents événements pour prendre cette menace au sérieux et pour la traiter au degré auquel elle doit l’être. À ce titre, les forces de sécurité intérieure ont déjoué treize attentats d’ultradroite depuis 2017. Je le rappelle ici, près de 1 300 personnes sont fichées S et, donc, suivies par nos services. l’occasion des récentes manifestations sauvages, nos forces de sécurité intérieure ont été largement mobilisées dans le cadre des enquêtes menant à l’interpellation de ces individus violents. C’est également ce gouvernement, monsieur le sénateur, qui a dissous, sur proposition du ministre de l’intérieur et des outre mer, de multiples associations ou groupements de fait s’inscrivant dans cette mouvance ultraviolente. Gérald Darmanin a pu d’ailleurs annoncer hier matin que trois autres groupuscules feraient l’objet d’une procédure de dissolution. Je parlais à l’instant de la Division Martel, dont le nom, vous le concéderez, nous donne une certaine idée du projet violent fantasmé par ces individus. Elle en fera partie. Monsieur le sénateur Brossat, les extrêmes, l’ultradroite, l’ultragauche –, sont des poisons pour notre démocratie. Ils doivent être combattus avec fermeté. C’est ce que nous faisons en remettant ces individus à la justice, en dissolvant des groupuscules tentés par l’ultraviolence contre nos concitoyens. La parole La parole est à Mme Anne Catherine Loisier, pour le groupe Union Centriste. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, dans la nuit de samedi à dimanche, des tirs en rafale se sont fait entendre dans le quartier Stalingrad à Dijon. Ces tirs d’armes de gros calibre sur un immeuble visaient non pas à intimider, mais à tuer. Les cibles étaient vraisemblablement de jeunes dealers, installés dans l’entrée, bien connue, de cet immeuble. Les jeunes ont pris la fuite sans être touchés, mais une balle a atteint un homme qui dormait, dans son lit, au premier étage.

de 57 % des homicides et tentatives d’homicide entre 2022 et 2023, face à l’ampleur des trafics qui gangrènent nos quartiers, mais aussi nos campagnes, quelles sont vos réponses ?

vous l’avez rappelé, dans la nuit de samedi à dimanche, un père de famille de 55 ans a été tué par balle dans son sommeil, à son domicile. J’ai une pensée sincère pour sa famille. Elle a perdu un proche, victime collatérale d’un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue. Lorsqu’un point de deal est particulièrement visé et harcelé par les services de police et de gendarmerie, comme celui de Dijon, nous le savons, les règlements de comptes et les batailles de territoire redoublent de violence. L’État ne reculera pas pour éradiquer le trafic de drogue. Le ministre de l’intérieur et des outre mer, Gérald Darmanin, a immédiatement envoyé et déployé la CRS 8 à Dijon. Ces renforts resteront autant de temps que nécessaire. Dans l’agglomération de Dijon, les services de l’État sont totalement mobilisés autour du préfet pour lutter pied à pied contre le trafic de stupéfiants, grâce au déploiement de moyens extrêmement importants. Depuis le début de l’année, dans le département de la Côte d’Or, 1 252 opérations ont été conduites, 2,4 tonnes 2,4 tonnes de stupéfiants saisies, 368 interpellations opérées. À l’échelon national, ce sont 14 410 opérations de démantèlement de points de deal qui ont été menées, en hausse de 30 % par rapport à 2022. Face au trafic de drogue qui gangrène nos quartiers, le Gouvernement déploie les moyens d’agir. Mais il faut aussi être intraitable à l’encontre des consommateurs. Car, sans consommateurs, je l’ai dit plusieurs fois, il n’y a pas de trafic, il n’y a pas de dealers. Madame la sénatrice, soyez assurée que le ministre de l’intérieur et des outre mer et l’ensemble du Gouvernement mettent tout en œuvre pour lutter efficacement contre ces fléaux que sont la délinquance et le trafic de stupéfiants. La parole

? Au delà d’une opération « coup de poing », la population de ces quartiers a besoin d’une présence dans la durée, pour s’assurer qu’elle ne se retrouvera pas seule face à ces bandes violentes. Quel dispositif le Gouvernement pense t il mettre en place en ce sens ?

plus dissuasives ? Enfin, nous le savons tous, la réponse pénale n’est pas à la hauteur de ce phénomène. Elle inquiète de plus en plus nos concitoyens, elle décourage les policiers et les gendarmes, elle nourrit le sentiment d’impunité chez les délinquants. La parole est à M. Yannick Jadot, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. Monsieur le président, avant de poser ma question, je tiens à rendre hommage à une infatigable écologiste, la députée européenne Michèle Rivasi, qui a disparu de manière aussi brutale que dramatique ce matin. Madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, demain débute la COP 28 à Dubaï, et c’est peu dire que les engagements climatiques des États sont insuffisants. Nous nous dirigeons vers un réchauffement planétaire de 3 degrés, soit deux fois plus que les engagements pris à Paris en 2015. « L’effondrement climatique a commencé

de gaz. Ce devrait être la seule boussole du président Macron à Dubaï et, madame la Première ministre, de votre gouvernement en France. À cet égard, comment allez vous empêcher le projet d’extraction du gaz de houille en Moselle ?

en taxant leurs superprofits,… Allez… … en supprimant toute aide publique, tout crédit d’impôt ou toute exonération de cotisations dont elles bénéficieraient. Monsieur le ministre, on ne mène pas la bataille du climat en signant des armistices avec les lobbys qui le détruisent. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour le groupe Les Républicains.

à Bruxelles, la présidence espagnole du Conseil de l’Union européenne. Voilà de quoi faire bondir nos concitoyens, en particulier nos agriculteurs, qui risquent une nouvelle fois d’être les dindons de la farce d’un processus politique qui dessaisit entièrement les parlements nationaux de leurs

La parole est à M. Frédéric Buval, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

en présence des acteurs institutionnels de chaque territoire ultramarin. En dépit de quelques malentendus regrettables, nous ne pouvons que saluer la volonté manifeste de coconstruction du Gouvernement. Pourtant, des inquiétudes demeurent, tant sur la forme que sur le fond.

en évaluer les conséquences et écouter les élus locaux pour prendre en compte les spécificités de chaque territoire et bâtir des solutions adaptées et différenciées.

des Ultramarins : ce que nous voulons, c’est une coconstruction productive. Le ministre chargé des outre mer recevra lundi 4 décembre l’ensemble des acteurs économiques ultramarins pour un point d’étape sur les mesures économiques prévues par le Ciom. Cette séquence de trois heures environ sera l’occasion pour chacun de poser des questions et de soumettre des propositions dans le cadre des réformes à venir, auxquelles les acteurs économiques seront bien évidemment associés. Par ailleurs, comme le ministre a eu l’occasion de le confirmer la semaine dernière, la réforme baisser les prix des produits de grande consommation, de garantir les ressources des collectivités et de protéger la production locale. Je le redis devant cette assemblée : aucune réforme n’est écrite Elle se fera en concertation avec les élus et le monde économique. À cet effet, les préfets constitueront dans les prochains jours des groupes de travail dans chaque territoire afin de recueillir des propositions. Le prochain bilan d’étape du Ciom, qui devrait se tenir à la fin du mois de février ou au début du mois de mars 2024, sera ainsi l’occasion de faire un point de situation sur les propositions formulées et de commencer à définir les premières modalités de cette réforme importante.

(CDPENAF) est une mesure de protection qui s’applique aux territoires à enjeux, autant dans l’Hexagone que dans les outre mer. Néanmoins, il est vrai que les territoires ultramarins sont intégralement

La parole est à Mme Jacqueline Eustache Brinio, pour le groupe Les Républicains.

D’un côté, une France qui a basculé dans une violence gratuite, une France où l’ivresse de la barbarie est le résultat d’une éducation défaillante et d’un refus d’accepter nos valeurs, une France « hors tout », souvent biberonnée à l’argent public ou vivant parfois de trafics, une France minoritaire certes, mais revendicative et omniprésente. De l’autre, une France paisible, respectueuse des lois, de l’autorité, une France civilisée qui aime s’amuser, s’instruire, s’engager, apprendre, une France tolérante, généreuse et ouverte d’esprit, qui subit quotidiennement l’autre France. Face à ce constat aussi désolant que préoccupant, nous méritons mieux que des leçons de morale ou des procès en stigmatisation ou en récupération politique. Les Français n’acceptent plus ce déni qui ne fait qu’accentuer davantage le fossé entre ces deux France. Vos litanies ne font qu’attiser les rancœurs et le sentiment d’injustice, et favorisent l’inquiétante envie de se faire justice. Face à face, nous y sommes ! Quand le Gouvernement écoutera t il enfin ceux qui n’ont qu’une seule volonté : l’unité de notre pays et la paix civile ?

on ne peut pas dire qu’il y aurait deux France qui s’opposeraient l’une à l’autre. Il y a, madame la sénatrice, une France : celle des villes, celle des champs, celle des cités, celle des cœurs de ville

il est ferme, et il est le même pour tout le monde. Aucun facteur potentiellement aggravant ne sera éludé ; rien ne sera caché. Je salue l’action déterminée des forces de police, notamment de la gendarmerie. Une mobilisation de 150 hommes a permis en moins de trois jours – ce qui est

Les morts de Samuel Paty, de Dominique Bernard, de Lola, d’Enzo et de Thomas sont des faits de société. C’est une réalité. L’impunité, le « en même temps » et votre aveuglement vous ont conduits à ignorer une France qui aspire clairement à l’autorité, à la fermeté et au respect ! Diriger, gouverner, c’est avoir du courage, de la cohérence. C’est ne pas céder aux minorités, c’est accepter d’écouter enfin cette majorité silencieuse qui n’en peut plus et qui ne veut plus subir Essentialiser les citoyens de ce pays, comme l’a fait le garde des sceaux hier, est inacceptable. Réveillez vous, tant qu’il en est encore temps

femme et ses enfants n’étaient plus protégées ni par une interdiction d’approcher ni par une ordonnance de protection. Les parents étaient en instance de divorce et avaient organisé une garde alternée. La mère s’est rendue deux fois au commissariat pour signaler des problèmes lors de la remise des enfants au père. Voilà…

Monsieur le président, madame la Première ministre, mes chers collègues, avant de prendre la parole pour la première fois dans cet hémicycle, je veux rendre hommage à mes prédécesseurs dans cette assemblée

Poadja. Chacun d’eux a défendu inlassablement le maintien de la Nouvelle Calédonie dans la République française. Mon action parmi vous s’inscrira dans cette même volonté : garder la Nouvelle Calédonie au sein de notre République de notre République ! Madame la Première ministre, la Nouvelle Calédonie, collectivité spécifique de la République, se trouve aujourd’hui à un carrefour décisif de son histoire. Le processus de décolonisation, encadré par les accords de Matignon et de Nouméa, a engagé la Nouvelle Calédonie sur la voie d’une autonomie accrue, respectueuse de son identité propre et de sa place unique au sein de la République. Le ministre de l’intérieur et des outre mer rentre tout juste de son cinquième déplacement en Nouvelle Calédonie. Je veux ici saluer l’engagement de votre gouvernement dans le dossier calédonien.

quand allez vous procéder au dégel du corps électoral pour les prochaines élections provinciales ? Les dizaines de milliers d’électeurs calédoniens exclus du corps électoral provincial veulent savoir quand et comment ils deviendront des citoyens calédoniens à part entière. Quand auront lieu les prochaines élections provinciales ? Ces élections sont capitales pour l’avenir de la Nouvelle Calédonie. Il est essentiel qu’elles soient organisées dans des conditions irréprochables afin d’assurer la légitimité du processus démocratique. La

vous l’avez rappelé, le processus politique prévu par l’accord de Nouméa a été mené à son terme et les Calédoniens ont choisi de rester français. Depuis plusieurs mois, le Président de la République et le Gouvernement s’emploient à organiser un dialogue serein et constructif avec les indépendantistes et les non indépendantistes. C’est la condition pour dessiner ensemble l’avenir de la Nouvelle Calédonie. Nous le devons à tous les Calédoniens, notamment à la jeunesse calédonienne qui a besoin de perspectives. Pour y parvenir, la méthode de mon gouvernement ne change pas. Nous voulons un dialogue avec toutes les parties prenantes, quelles que soient leurs convictions. La main de l’État est toujours tendue, y compris à ceux qui, parfois, s’éloignent de la table des discussions. Nos objectifs, eux non plus, ne changent pas. Nous voulons parvenir à un accord sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle Calédonie. Le Gouvernement a émis des propositions qui servent de base aux discussions. Néanmoins, les prochaines élections provinciales devront avoir lieu avec un corps électoral dégelé. C’est une exigence démocratique, comme l’a rappelé le ministre de l’intérieur et des outre mer Gérald Darmanin lors de son déplacement en Nouvelle Calédonie la semaine dernière. Les discussions doivent donc se poursuivre pour parvenir, je l’espère, à un accord politique. Mais dans le même temps, le Gouvernement avance. Le Conseil d’État a été saisi pour préciser les conditions juridiques d’évolution des règles en matière électorale. nous proposerons les textes nécessaires au dégel du corps électoral et au report des élections provinciales. Quoi qu’il en soit, ces élections se tiendront en 2024. Monsieur le sénateur, avec mon gouvernement, nous cherchons un accord global sur le dégel du corps électoral, bien sûr, mais aussi sur la citoyenneté calédonienne, l’autodétermination, le statut et les institutions. Dans ce contexte, je compte sur l’esprit de responsabilité de chacun pour que les discussions soient menées dans un esprit d’ouverture. Il y va de l’avenir de la Nouvelle Calédonie. La parole

Guidez, pour le groupe Union Centriste. Ma question s’adresse à Mme la ministre des solidarités et des familles. L’annonce de l’adoption d’une loi Grand Âge avant la fin 2024 est une bonne nouvelle. Il est urgent de tenir les engagements pris pour s’occuper dignement des personnes âgées vulnérables et des professionnels qui les accompagnent. Pour répondre aux besoins de nos aînés, il est indispensable de financer le ratio de huit professionnels pour dix personnes âgées en établissement, ainsi que ce devrait être le cas depuis 2012 et comme le préconisent la Défenseure des droits, la Cour des comptes et le Haut Conseil de la

Les récentes enquêtes sont préoccupantes et alertent sur des difficultés d’une ampleur inédite. La survie de certains établissements et services est en jeu. Face à la gravité de la situation, il est nécessaire de prendre des mesures fortes et de long terme pour éviter la faillite de certains établissements et services, acteurs indispensables de l’accompagnement des personnes âgées. la ministre, comptez vous répondre à cette situation d’urgence au travers d’une loi pluriannuelle pour le grand âge ? Si oui, quand, comment et avec quelles mesures concrètes ? Quels sont les contours de votre plan Grand Âge et autonomie ? Nous espérons une réponse engagée. La parole

En effet, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique avait été adoptée par le Parlement, notamment avec l’aide des députés européens Renaissance, cette même consigne dont nous avions eu collectivement la sagesse de repousser la mise en œuvre, cette même consigne à laquelle vous, ministre de la transition écologique, vous êtes opposé de manière éloquente, reprenant au demeurant point par point les arguments de notre rapport d’information relatif Peut être faut il chercher l’origine de ce soutien du côté de l’Élysée ? Le Président de la République semble avoir fait de la consigne pour recyclage le nouvel avatar de son marketing écologique.

un dispositif de préfiguration de consignes régionales, si certains territoires qui sont très en retard décidaient de combler leur retard de cette manière. Je rappelle en effet que, derrière les statistiques nationales,

samedi dernier dans la presse sur le rôle déterminant joué par l’immigration dans la prospérité économique de notre pays. Dans les dix années à venir, la France aura « sans doute besoin d’avoir recours à l’immigration », a t il déclaré, car 1,3 million d’emplois seront à pourvoir rien que dans le secteur de l’industrie, du fait des départs à la retraite. 100 000 et 200 000 personnes venant de l’étranger pourraient être nécessaires pour réindustrialiser notre pays – et, encore, c’est une estimation basse. Il faudrait en effet dans le même temps que notre pays soit capable de former dans ce secteur « 800 000 à 900 000 jeunes et moins jeunes ». Ma question est simple : comment le Gouvernement

Vous savez, le projet de loi Immigration que défend le Gouvernement est actuellement examiné par la commission des lois à l’Assemblée nationale, après avoir été voté ici au Sénat. Le Gouvernement reste attaché à ce que les étrangers qui contribuent à la vitalité de notre économie et de notre pays puissent être régularisés, selon des modalités qui doivent encore être définies au cours des discussions à venir, notamment parlementaires, particulièrement dans les secteurs en tension. Les étrangers vivent et travaillent parfois depuis très longtemps en France sous l’autorité de patrons qui peuvent refuser de les régulariser. Nous souhaitons mettre fin à ce servage moderne, en permettant ces régularisations grâce à ce projet de loi. Comme vous, nous sommes en effet convaincus que le travail demeure un facteur d’intégration puissant des étrangers primo arrivants. Il est de notre devoir de garantir les meilleures conditions d’intégration à celles et à ceux qui ont notamment obtenu l’asile dans notre pays.

En effet, l’examen du projet de loi Immigration Intégration aurait dû faire émerger une vision stratégique et globale. Oui, la France aura un besoin impératif de travailleurs étrangers, au risque de connaître une régression économique majeure qui dégradera notre prospérité, notre attractivité et notre influence.

Agents de sécurité, médecins hospitaliers, aides soignantes, vétérinaires, emplois agricoles : cette France qui se lève tôt, voire très tôt, contribue à la richesse nationale. Quand d’autres pays européens font le choix d’une politique volontairement intégratrice, le projet de loi pour contrôler l’immigration prépare le déclassement économique de notre pays. Il est examiné à l’Assemblée nationale aujourd’hui, il est encore temps de rectifier le tir.

Un don en direct à des associations aurait permis à l’acheteur du ticket de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % et de véritablement accompagner celles ci. Au delà des aspects financiers, la question de l’addiction est centrale.

Comment l’État peut il participer directement et aussi cyniquement à ce scandale sanitaire ? Comment le Président de la République a t il pu s’ériger en VRP de la Française des jeux le week end dernier dans le Jura ? Verrons nous demain la création par le Gouvernement de nouveaux jeux de loto pour pallier les carences des politiques publiques ? Je vous suggère dans ce cas le loto du handicap, le loto du grand âge, le loto des maladies rares, le loto des soins palliatifs et, à terme, pourquoi pas, le loto de la prévention des addictions, notamment aux jeux ! Pourquoi

La parole est à M. Jean Jacques Panunzi, pour le groupe Les Républicains.

Notre île connaît cette maladie depuis 2001, mais c’est la première fois qu’elle est confrontée au variant 8, particulièrement virulent. Lorsque l’on regarde la carte des sérotypes en Europe, on s’aperçoit que le variant qui touche aujourd’hui la Corse n’existe qu’en France continentale. Il y a donc une double faille dans le processus

Quand une partie du cheptel est décimée, on ne peut le renouveler facilement par achat. Pour maintenir l’AOP, il faut miser sur la reproduction ; le parcours est long et semé d’embûches. et semé d’embûches. Si la prise en charge du vaccin a été réglée par les services préfectoraux et la collectivité de Corse, l’indemnisation des animaux morts ou atteints de morbidités reste en suspens. la souveraineté alimentaire en Corse sont bien en deçà des besoins en pleine épidémie. On ne peut pas raisonner à enveloppe fermée, tout simplement parce que l’on ne connaît pas encore l’étendue des dégâts

La seule voie d’indemnisation possible est celle du règlement général d’exemption par catégorie, qui permet aux États membres d’octroyer des aides, après notification à Bruxelles bien sûr, pour faire face à des impondérables.

est une maladie virale qui touche les ruminants sauvages et domestiques, les ovins, les bovins et même les caprins. Elle a touché à plusieurs reprises le territoire national ces dix dernières années. Elle est strictement animale, elle n’affecte pas l’homme, elle n’a aucune incidence sur la qualité sanitaire des denrées, que ce soit la viande ou le lait. Toutefois, vous l’avez souligné, ces répercussions économiques peuvent être importantes, directement, parce que les animaux infectés peuvent présenter des signes cliniques ou, indirectement, par la fermeture de marchés étrangers. De nombreux foyers cliniques de fièvre catarrhale ovine de sérotype 8 sont constatés dans des élevages depuis le début du mois d’août dernier sur le territoire métropolitain. Plus de 1 630 foyers sont aujourd’hui recensés, notamment dans l’Aveyron, La vaccination est un outil de prévention et de lutte qui permet de protéger le cheptel et son voisinage. Elle est volontaire. L’éleveur peut vacciner directement ses animaux. En revanche, si elle doit être justifiée et certifiée, la vaccination doit alors être réalisée par un vétérinaire. La réglementation européenne prévoit que les mesures de prévention et de lutte relèvent de la responsabilité de la profession agricole. C’est pourquoi l’État n’a généralement pas vocation à prendre en charge le coût de la vaccination ni à indemniser les pertes économiques induites par cette maladie. Les organisations professionnelles agricoles se sont organisées rapidement pour établir un document de recommandation aux éleveurs. L’introduction du virus en Corse est particulièrement récente. On recense actuellement une vingtaine de foyers confirmés de sérotype 8, 3 et 4.

Monsieur le président, madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l’explosion de l’insécurité que connaît la France, si dramatique soit elle, ne doit pas nous détourner de la catastrophe économique et sociale que nous traversons. À cet égard, la litanie statistique est éloquente. 32 % des Français ne sont pas en mesure de se procurer une alimentation saine et en qualité suffisante pour manger trois repas par jour ; 15 % sautent des repas ; 43 % déclarent avoir des difficultés pour manger des fruits et légumes frais quotidiennement.

Avec un taux de pauvreté de la population française de 15 %, soit 10 millions de personnes, le bilan du Gouvernement est catastrophique. Qui plus est, alors que le froid arrive, 44 % des Français disent se priver de chauffage. Quand on a de l’argent, on fait des choix ; quand on n’en a plus, on fait des sacrifices. on fait des sacrifices. Mon discours n’est pas misérabiliste, il n’est que le reflet de ce que vivent les Français. Rien ne s’améliore, tout s’aggrave et aucune des politiques que mène ce gouvernement n’inverse la tendance, car tout n’est que cataplasme quand c’est d’un changement profond de système que nous avons besoin. Le Gouvernement pèche par orgueil en refusant de voir la réalité du drame économique et social que nous vivons et du déclassement français que nous connaissons. On va me répondre, comme d’habitude, que les causes de ce marasme sont conjoncturelles. Pour notre part, nous pensons qu’elles sont aussi structurelles. La crise sanitaire et les conflits internationaux ne peuvent pas être une éternelle réponse à tout.

ni celui de l’opération du Saint Esprit. C’est parce que le Gouvernement a veillé à réduire les dépenses contraintes et à relever les revenus, en particulier les petits revenus.

la proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP, de la proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques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

la taxe foncière de l’une peut être jusqu’à cent fois plus élevé que celui de l’autre. Cette différence de traitement met en danger l’équilibre économique de certaines centrales en ombrière déjà installées et compromet le développement de ce type de projet.

à Mme Jocelyne Guidez. Le présent amendement tend à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les maisons de santé financées par les professionnels de santé qui y travaillent. Ces établissements sont pluriprofessionnels : des professionnels médicaux, des auxiliaires médicaux, des pharmaciens ayant acquis ou louant les locaux y exercent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours.

à une rupture d’égalité entre deux types de structures ayant le même objet ; les professionnels libéraux exerçant dans des structures mises en place par des collectivités locales bénéficient de conditions d’exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées. Pourtant, ceux ci sont soumis aux mêmes obligations d’accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires. Quel

d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il vise ainsi à établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB.

des contraintes et une déontologie, en matière académique notamment. Je

dans un contexte de raréfaction du foncier et alors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge, sans délai, par la collectivité concernée, il paraît justifié de permettre aux collectivités locales de supprimer ce plancher de 40 vestige de la part départementale de la taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme cela était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.

L’objectif est de mobiliser les particuliers aux côtés des investisseurs institutionnels afin de répondre aux besoins croissants de logements. Cet amendement vise à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant dix ans, les nouveaux logements acquis en l’état de futur achèvement et destinés à la location nue à usage d’habitation principale. Cette exonération est conditionnée par un engagement de location du bien d’une durée minimale de dix ans. Cette proposition ne vise pas à introduire un nouveau dispositif fiscal, il s’appuie sur le régime existant de loueur meublé non professionnel, créé en 1948. Elle vise à activer une source de financement complémentaire pour le logement locatif intermédiaire, qui est crucial pour la cohésion sociale dans les zones soumises à des tensions immobilières.

et de l’habitation. Or, dans les faits, cette autorisation n’est délivrée, la plupart du temps, qu’une fois que tous les logements sont vides. Elle intervient donc à la fin d’une procédure qui peut durer plusieurs années, le temps de reloger tous les locataires. Cette situation conduit souvent, en pratique, à priver d’effet la mesure de dégrèvement, puisque les organismes d’HLM doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir. C’est pourquoi il est proposé ici de faire référence, non pas à l’autorisation définitive de démolir, mais à la décision du préfet de « prise en considération du dossier d’intention de démolir ». Par cette décision, le préfet prévaliderait la demande d’autorisation de démolir après avoir vérifié le respect de la réglementation, la justification du projet et l’accord des autorités locales.

à raison de la propriété d’un bien. Il doit demeurer d’une application stricte et précise. Les règles en vigueur lient l’octroi du dégrèvement à une autorisation garantissant la réalisation de l’opération. Le simple dépôt d’une demande n’apporterait pas cette assurance et fragiliserait juridiquement l’application du dégrèvement. Il existe un risque de fraude manifeste. La disposition que vous proposez poserait de grandes difficultés au service du contrôle fiscal. J’y suis donc défavorable.

exonération de taxe foncière pour les propriétaires qui confieraient la gestion de leurs parcelles à des groupements forestiers. Autrement dit, nous encourageons le regroupement foncier des parcelles afin de favoriser une gestion plus durable et cohérente de nos forêts. L’amendement

réalisées pour un motif sanitaire. En outre, l’exonération de taxe foncière serait réservée à la plantation d’essences diversifiées afin de décourager la monoculture et d’inciter aux travaux d’ensemencement ou de plantation vertueux.

des activités annexes en complément de leur activité principale. Cette diversification, observée au sein des exploitations, est un levier essentiel de la pérennité financière du monde agricole de l’île. Cet amendement de M. Parigi vise donc à sécuriser les exploitants agricoles corses en exonérant de la taxe foncière les bâtiments agricoles à usage mixte, quelle que soit la surface du bâti consacrée à d’autres activités non agricoles.

a adopté l’alignement de l’exonération de la taxe d’habitation pour les établissements sanitaires, sociaux et médico sociaux privés non lucratifs,

les propriétaires de locaux d’habitation déclarent, à compter de 2023, l’interface numérique Gérer mes biens immobiliers du site impots.gouv.fr, le statut d’occupation et l’occupant des logements qu’ils détiennent. Ils déclareront aussi prochainement le loyer acquitté par les locataires, ce qui donnera aux services fiscaux une image fidèle et exhaustive du marché immobilier, indispensable pour engager la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.

par l’article 103 de la loi de finances initiale pour 2023. Il est donc proposé de faire évoluer la collecte des loyers des locaux professionnels en capitalisant sur l’interface

plus fiable que les déclarations actuellement prévues par le mode d’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels. Enfin, cet amendement tend à supprimer la section IV, « Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants pour replacer l’article 1418 dans sa section originelle, « Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d’habitation ». Très bien

a prévu de déterminer des coefficients d’actualisation des valeurs locatives pour les locaux professionnels. Ceux qui, comme moi, ont participé aux travaux des

disposer d’une année supplémentaire pour intégrer les résultats des travaux d’actualisation dans les bases d’imposition dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. C’est précisément la décision qui a été prise en concertation

n° I 368 rectifié. La loi de finances pour 2020 a prévu que la valeur locative des locaux d’habitation à caractère exceptionnel serait calculée en appliquant un taux de 8

arbitraire parce que le principe d’une rentabilité de 8 % ne repose sur aucune réalité économique. C’est sans compter que ces biens sont souvent situés en zone rurale, où la demande locative de bâtiments de grande taille n’existe pas. Il est excessif encore parce que les charges qui pèsent sur ces immeubles sont des sources de coûts et non de profits, alors que le bâti traditionnel rapporte rarement plus de 4 %.

que nous avons défendus en loi de finances pour 2022. Nous avons organisé une collecte spécifique des données relatives aux locaux d’habitation ayant des caractéristiques exceptionnelles. Ainsi,

Un EPCI créé par fusion à compter du 1 janvier 2018 est contraint de continuer à verser aux communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle, dans le cadre de leurs attributions de compensation, la contrepartie prévue dans code général des impôts sans plus bénéficier de la recette de la taxe d’habitation qui justifiait ce versement puisqu’elle n’est pas intégrée au calcul de la compensation de TVA perçue par l’EPCI issu de la fusion dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation.

Il est cohérent avec les engagements du Gouvernement d’une compensation à l’euro près de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les collectivités. Il y a un an, le Sénat avait déjà débattu de cet amendement, qui avait reçu un avis favorable et avait été voté. Le Gouvernement Le Gouvernement s’était engagé à régler ce problème dans l’année. Malheureusement, un an après, rien n’a été fait ; la situation est toujours la même. Cet amendement vise donc à régler cette situation.

l’avis du Gouvernement ? Les modalités de compensation que vous souhaitez faire évoluer ont été validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 octobre 2022. Par conséquent, l’avis est défavorable.

De la même manière, elles ne s’appliquent pas aux communes qui ont intégré le taux additionnel de taxe d’habitation à leur taux communal après avoir quitté un syndicat bénéficiant d’une contribution fiscalisée. Aussi, le présent amendement vise à prévoir, dans l’esprit des dérogations déjà accordées par le législateur, qu’une exception puisse être également appliquée aux communes ayant augmenté ce taux à la suite d’un changement d’EPCI à fiscalité propre ou d’un retrait d’un syndicat, intervenu entre 2017 et 2019. L’amendement n° I 1039 rectifié,

Selon l’article 1609 du code général des impôts, cette possibilité est aujourd’hui réservée aux seuls syndicats mixtes composés exclusivement de communes ou aux syndicats mixtes composés de communes et d’EPCI, et d’EPCI, en remplacement de la contribution budgétaire des communes ou des communautés de communes associées. Il s’agit donc d’étendre cette possibilité à d’autres types de syndicats mixtes.

d’EPCI, instauré par la loi de finances de 2010, ne s’appliquant pas aux situations de changement de régime fiscal à périmètre constant. En conséquence, le dispositif de droit commun basé sur l’instauration d’une Tascom communautaire et l’application d’un coefficient minimum s’applique la première année.

parallèle, de nombreux contribuables enregistrent une fluctuation anormale de leurs cotisations : une baisse la première année, puis une augmentation jusqu’au niveau antérieur, voire au delà, selon les coefficients précédemment votés.

Toutefois, elle reste encore peu utilisée aujourd’hui, en particulier en raison de l’impossibilité, à ce jour, de la sectoriser. De fait, toutes les friches commerciales ne sont pas porteuses des mêmes enjeux fonciers ; ainsi, de nombreuses communes et EPCI à fiscalité propre souhaitent cibler cette taxe sur les sites destinés à une reconversion, ce qui n’est pas possible aujourd’hui.

vise donc à faciliter le recours à cet outil fiscal en autorisant son instauration dans certains secteurs, sur décision de la collectivité concernée. Le conseil municipal ou communautaire serait ainsi conduit à en motiver le périmètre eu égard à l’importance des opérations d’aménagement ou de requalification en cours ou à venir ou aux travaux substantiels de voirie, de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain,

Mme Isabelle Briquet. que la plupart de nos concitoyens rencontrent des difficultés pour se loger, il est difficilement acceptable que la fiscalité du logement ne soit pas adaptée aux revenus des particuliers. Actuellement, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683 est fixé à 3,8 %. Il peut être modulé par les conseils départementaux, mais indépendamment de la valeur du bien.

en raison du retournement du marché immobilier. On constate ainsi une baisse moyenne de près de 23 % de ces droits entre septembre 2022 et septembre 2023.

volatilité de cette recette majeure pour les départements pourrait donc être atténuée par la légère majoration du taux sur les transactions de luxe que nous proposons.

insupportable et intolérable.

d’hébergement d’urgence et de solutions de relogement temporaire dans le secteur social, d’une part, et de l’existence de foncier vacant, d’autre part, de nouvelles solutions de construction durables, déplaçables, démontables et réemployables ont vocation à apparaître sur tout le territoire. vise à introduire un dispositif d’exonération de taxe d’aménagement et de taxe d’archéologie préventive en faveur de ce nouveau type de constructions. En mobilisant des sites inoccupés ou en attente d’affectation, les constructions déplaçables permettent de répondre non seulement à la demande de relogement provisoire, mais aussi aux enjeux de la ville durable en termes de construction et de performance environnementale des bâtiments, de réemploi des ressources, d’inclusion sociale et de rénovation urbaine. Cet amendement tend donc à étendre le champ d’application du taux réduit de TVA pour encourager le développement de ce type de constructions durables et réemployables, destinées au relogement provisoire des habitants du parc social et à l’hébergement des publics précaires, en établissant un cadre fiscal favorable.

sénateur, le taux réduit de TVA à 5,5 % est déjà applicable aux livraisons de locaux à usage des structures du secteur social et médico social visés par la mesure.

Aujourd’hui, seulement 6 millions de Français, soit un Français sur dix, contribuent au service de gestion et de traitement des déchets une tarification incitative. Si cette argumentation n’emporte pas votre adhésion, monsieur le rapporteur général, il

Le plafond de cette taxe, qui a été réduit de 3 euros à 1,50 euro par la loi de finances pour 2007, n’a pas été réévalué depuis. Or la majorité des taxes et impôts ne sont pas plafonnés.

doivent pouvoir, si elles le souhaitent, augmenter le montant de cette taxe. J’ajoute que cet amendement a été adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi de finances pour 2023, puis supprimé par l’Assemblée nationale. La parole

Martine Berthet. Depuis le dernier renouvellement des baux de pêche fluviaux et lacustres de l’État pour la période 2017 2021, l’autorisation d’amarrage et de stationnement des bateaux de pêche n’est attribuée aux pêcheurs professionnels que moyennant le paiement de la redevance prévue à l’article L. 2125 1 du code général de la propriété des personnes publiques. Or contrairement aux autres navigants professionnels du domaine public, les pêcheurs professionnels paient déjà un droit d’occupation de ce domaine, sous forme de loyers, les autorisant à amarrer et à stationner leurs embarcations, à naviguer et à exercer une activité économique. Afin de remédier à cette difficulté, l’article 172 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 devait permettre aux pêcheurs professionnels de pouvoir continuer à occuper le domaine public sans paiement supplémentaire pour la délivrance de l’autorisation d’occupation

en eau douce puissent bénéficier de la gratuité systématique pour la délivrance de l’AOT. Quel

à M. Dominique Théophile. L’article 78 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé en Guadeloupe et en Martinique un régime expérimental de vente hors taxes au bénéfice des croisiéristes qui y font escale. Ce dispositif, que j’avais défendu dans cette assemblée, vise à renforcer la compétitivité des territoires dans lesquels il s’applique par le biais du développement du commerce local. Créé pour une durée de quatre ans initialement, il n’est toujours pas entré en vigueur, en raison principalement de la crise du

pour les BRS conclus avec un opérateur chargé de vendre les droits réels immobiliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble des livraisons et livraisons à soi même et, sur délibération des communes et de leurs groupements, un abattement de la taxe foncière sur les

Malgré la difficulté croissante pour les ménages, notamment pour les plus modestes, d’obtenir des prêts bancaires, la propriété reste un objectif attractif pour de nombreux Français, d’autant que le marché locatif ne peut absorber la forte augmentation de la demande à lui seul. En 2015, le bail réel solidaire a été mis en place pour permettre de développer une offre de logements en accession sociale pérenne. Ce dispositif permet à des ménages d’accéder à la propriété à des

Afin d’éviter cette situation, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les organismes de foncier solidaire au droit fixe de 125 euros, la cession des droits aux ménages restant, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles de droit commun.

au développement de ce type de constructions durables et réemployables, destinées au relogement provisoire des habitants du parc social et à l’hébergement des publics précaires. Quel est l’avis de

ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales qui ont bénéficié du produit des DMTO issus de l’acquisition. Or il peut y avoir un délai de plusieurs années entre le versement du dégrèvement par les collectivités et la restitution des DMTO à la suite de l’acquisition.

L’objet de cet amendement est clair : dans un contexte de rareté des fonds publics, il n’est plus admissible d’allouer des montants substantiels d’argent public aux entreprises sans contrepartie ni considération pour l’intérêt général. Notre proposition cible spécifiquement les entreprises assujetties à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière, catégorie englobant au minimum les sociétés cotées de plus de 500 salariés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros ainsi que les sociétés non cotées dépassant les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Tout l’intérêt de cet amendement réside dans son approche systémique : il s’agit d’étendre la conditionnalité à toutes les formes d’aide publique, y compris les subventions, les garanties de prêt, les garanties publiques pour le commerce extérieur, l’éligibilité aux crédits d’impôt, et ainsi de suite. Les standards qui devront être respectés par les entreprises concernent des domaines cruciaux tels que la réduction de gaz à effet de serre, le contrôle des licenciements à caractère spéculatif, l’encadrement des écarts de salaire, l’interdiction de versement de dividendes sans bonification de salaire, la lutte contre les discriminations, le devoir de vigilance et l’interdiction de la détention d’actifs dans des paradis fiscaux. Pour garantir l’applicabilité de cette mesure, des pénalités financières sont prévues en cas de non respect des obligations définies. En adoptant cet amendement, le Sénat enverrait un signal fort. Les aides publiques doivent être alignées sur les valeurs de responsabilité sociale et environnementale que nous défendons et que les entreprises mettent beaucoup en avant dans leur communication.

M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

autres que les collectivités territoriales, leurs groupements et les administrations de sécurité sociale. Le total de la fiscalité affectée s’élève pour 2024 à plus de 360 milliards d’euros, dont 231 milliards d’euros pour les organismes de sécurité sociale, 56 milliards d’euros pour le secteur local et plus de 44 milliards d’euros pour les organismes divers d’administration locale. Le montant de cette fiscalité affectée est même supérieur au produit des recettes fiscales nettes de l’État

Merci